la diffusion, la révélation et la transmission de données identifiantes ou permettant la localisation d'une personne, quelle qu'elle soit, avec un quantum de peines renforcé lorsque ces faits visent une certaine catégorie de personnes. La rédaction initiale de l'article 24 visait effectivement un cas particulier de ce cas général, en ayant pour objet la diffusion d'images ou de données identifiantes. Toutefois, la rédaction du Sénat, adoptée en commission mixte paritaire, ne fait plus de l'article 24 un cas particulier de l'article 18. En effet, elle crée une infraction dont le libellé montre qu'elle est sans lien avec la diffusion de données. données. La provocation à l'identification peut s'opérer sans diffusion de données. Les deux infractions ne visent donc plus la même chose : soit il y a provocation à l'identification pour les catégories de personnes visées par l'article 24, à savoir les policiers, les gendarmes et les douaniers en opération, et celui-ci s'applique, qu'il y ait ou non diffusion de données identifiantes ; soit, toujours dans le cas restreint des personnes visées à l'article 24, il y a diffusion de données identifiantes sans provocation, et l'article 18 s'applique. La question pourrait éventuellement se poser dans les cas où il n'y a pas de provocation explicite. Dans les exemples donnés par le ministre de l'intérieur et le directeur général de la police nationale, il s'agit de la diffusion de photos sur un site sans autre mention. La provocation implicite n'existe pas, c'est la raison pour laquelle la deuxième partie de l'article 24, dans la rédaction du Sénat issue de la commission mixte paritaire, réprime la constitution de fichiers destinée à nuire. Quand quelqu'un cherchera à nuire aux forces de l'ordre par l'identification des agents en opération, s'il appelle à les identifier ou s'il constitue des fichiers, il tombera sous le coup de l'article 24 ; s'il diffuse leurs identités, adresses ou localisations sans rien dire de plus,

sachant, hélas, dans cette matière comme dans d'autres, que l'on ne peut pas réécrire l'histoire. Voilà, c'est ainsi qu'est né l'article 18. De la même façon, entendez, monsieur le sénateur, que je sois blessé à l'idée que vous considériez que la liberté de la presse est votre monopole. Vous avez commencé fort, vous aussi,

contre un méchant ministre voulant la museler. Il faut être sérieux, à un moment donné ! L'article 18 ne concerne en rien les journalistes. Il vise les gens qui propagent la haine

Nous travaillons de manière austère et très impliquée depuis plusieurs jours et plusieurs nuits. Je souhaiterais, indépendamment de l'animosité que le garde des sceaux peut ressentir à l'égard de tel ou tel, ... Mais je ne vous connaissais pas qu'il soit possible, en tant que parlementaire, d'intervenir ici sans que soient utilisés des qualificatifs grossiers ou insultants.

vote. Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, il y a des caricatures qui ne sont pas conformes à la réalité. Depuis plusieurs semaines, Mme Marie-Pierre de La Gontrie met l'accent sur les problèmes de compatibilité entre l'article 24 de la précédente loi et l'article et l'article 18 du présent texte. C'est un débat de fond. À cet égard, monsieur le garde des sceaux, je voulais vous dire- très calmement, vous le voyez -que notre groupe a beaucoup réfléchi sur cet article 18. Moi aussi ! La vie privée des journalistes mis en cause est une vraie question. Vous aurez sans doute observé, monsieur le garde des sceaux, que notre groupe n'a pas proposé de supprimer l'article 18. Nous avons simplement déposé un amendement de

des débats outranciers ; il y a lieu simplement d'examiner les textes, ainsi que notre position, qui n'est en rien caricaturale.

pour le monde du journalisme comme pour la compatibilité des deux articles. Je

ces révélations ne sont pas nécessairement le fait de journalistes. La loi de 1881 protège, au-delà des journalistes, la liberté d'expression. Il n'empêche que,

vous proposons d'insérer : « Cette disposition n'a pas pour objet et ne peut avoir pour effet de réprimer la révélation ou la diffusion de faits, de messages, de données, de sons ou d'images qui ont pour but d'informer le public alors même que ces informations pourraient ensuite être reprises et retransmises par des tiers dans le but de nuire à la personne qu'elles permettent d'identifier

le nouveau délit n'a pas pour objet de réprimer la diffusion de propos, sons ou images ayant pour objet d'informer le public- c'est le travail des journalistes -, quand bien même ces informations seraient utilisées par des tiers dans le but de nuire. L'équilibre du dispositif répressif au regard de la liberté d'expression et de la communication réside dans l'existence d'un élément intentionnel spécifique permettant de réserver l'application du délit aux seules personnes ayant intention de nuire. Madame la rapporteure,

alors que cette garantie n'est prévue que pour certains délits de presse ? Oui ? Non ? Pas de réponse. Troisièmement, la détention provisoire, qui est possible

dans le code de procédure pénale la possibilité d'extraire les haineux, qui n'ont rien à faire dans la loi de 1881 et qui viennent s'y lover, pour faire en sorte que ceux-ci soient immédiatement jugés.

la loi pénale ne doit effectivement pas se permettre d'être floue. Si la loi du 29 juillet 1881 est d'une complexité sans nom, elle est tout de même précise.

: s'agissant des personnes visées alors, elle a redéfini qui devait rester sous l'empire de la loi de 1881. Ce faisant,

Je ne comprends pas pourquoi vous vous êtes opposé à ce que cette précision, très importante pour nous, figurât dans le texte. Pour nous,

quant aux condamnations de personnalités pour crimes ou délits. En fait, cela donne aux juges le pouvoir de prononcer ce qui s'apparente à une peine complémentaire. Nous voulons instituer une véritable peine de diffusion à la télévision de ces condamnations. Quel est l'avis de la commission ?

Madame la sénatrice de La Gontrie, vous êtes cordialement invitée à la Chancellerie. Franchissez-en donc la porte, venez me parler de cette difficulté : vous verrez que nous pourrons travailler ensemble.

adjoindre la situation du non-lieu ou du classement sans suite dans le texte, pour permettre aux personnes de se défendre dans tous les cas de figure.

Il faut lutter contre les sites miroirs reprenant des contenus jugés illégaux par l'autorité judiciaire, gardienne des libertés fondamentales, afin de prévenir plus efficacement la réapparition de tels contenus. Il est nécessaire de mettre en place une procédure pour assurer l'effectivité d'une décision de justice constatant l'illicéité d'un site internet et ordonnant son blocage ou son déréférencement, en permettant d'ordonner judiciairement le blocage de sites dédiés à la diffusion de contenus illicites. Nous Nous pouvons d'ailleurs saluer le rétablissement de la place du juge dans le dispositif prévu à cet effet, à la suite du vote du texte par l'Assemblée nationale. Toutefois, un véritable problème demeure. Le constat de la similitude entre les contenus du site et du site miroir est laissé à la libre appréciation de l'autorité administrative. De plus, le critère proposé par l'article- avoir un contenu « identique ou équivalent » -manque tout de même de précision. Ne reposant pas sur le caractère manifeste de la similitude, les décisions pourraient être prises arbitrairement, voire conduire à des atteintes disproportionnées à la liberté d'expression.

contenu. La majorité sénatoriale n'a pas pris ce parti

article, qui se contente de rappeler des dispositions déjà existantes, sans rendre obligatoire aucune mesure, risque d'être totalement inefficace dans la lutte contre la propagation de contenus haineux sur internet. Notre demande de suppression de cet article s'explique donc par l'inefficience

miroirs. Le projet de loi permet désormais à l'administration de demander aux intermédiaires techniques, fournisseurs d'accès à internet et hébergeurs de bloquer l'accès à ces sites, de les déréférencer des moteurs de recherche et de les inscrire sur une liste noire à destination des annonceurs publicitaires. Lorsque la justice

de temporalité que je souhaite rappeler. Le texte européen a été présenté le 15 décembre 2020, alors même que le projet de loi a été présenté le 8 ou le 9 décembre 2020. La France

la proposition de loi sur les contenus haineux. Un certain nombre de sites illégaux font l'objet d'un blocage par la justice française. Le processus est toujours le même : il faut plusieurs mois à la justice pour bloquer le site-

Selon une jurisprudence du Conseil constitutionnel, dès lors que les surcoûts sont importants, ils doivent être pris en charge par l'État. Mais le Conseil d'État a indiqué que si les surcoûts étaient négligeables, ils pouvaient être laissés à la charge des FAI, des hébergeurs ou des autres intermédiaires techniques.

qui contreviennent à la loi sur internet ? Nous ne pourrions pas le faire même si nous avions 2 500 magistrats affectés uniquement à cette tâche

nationale avait doublement étendu la notion de site miroir, en mentionnant les contenus équivalant à tout ou partie du contenu du service visé par une précédente décision de justice, et non plus seulement les contenus reprenant en totalité ou de manière substantielle le contenu du service visé par la décision de justice. La commission des lois du Sénat a souhaité, utilement, circonscrire le champ d'application de cette disposition. Cependant, en prévoyant que l'autorité administrative ne peut apprécier de manière autonome le contenu des sites en question, il nous semble qu'elle est peut-être allée un peu trop loin

est à Mme Sabine Drexler. Cet amendement de ma collègue Valérie Boyer vise à étendre les dispositions de la lutte contre la haine en ligne, en ajoutant à l'apologie des crimes contre l'humanité la négation et la banalisation des crimes de génocide. Cette disposition imposerait notamment aux plateformes de lutter contre la diffusion de contenus niant le génocide arménien en ligne, dont la pénalisation reste inconstitutionnelle à ce jour. En 1990, le législateur a fait du négationnisme un délit de presse. En adoptant la loi Gayssot, il interdisait de contester publiquement un ou plusieurs crimes contre l'humanité « tels que définis par le statut du tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945 Conçue à l'origine comme une limite à la liberté d'expression, cette réponse pénale au mal irrationnel qu'est l'antisémitisme s'est cherchée pendant vingt-cinq ans, au gré des combats et inquiétudes de toutes parts. D'un côté, les rescapés de la Shoah qui, après avoir vécu l'invivable, comble du vice, que leur calvaire n'avait jamais eu lieu. De l'autre, les historiens et chercheurs- ceux de bonne foi -qui s'inquiétaient d'être traînés en correctionnelle pour avoir exercé leur métier. Le 29 mai 1998, l'Assemblée nationale adoptait le principe, selon lequel « la France reconnaît publiquement le génocide arménien de 1915 ». Ce principe devenait officiellement une loi de la République avec la loi du 29 janvier 2001 relative à la reconnaissance du génocide arménien de 1915. En reconnaissant l'existence du premier génocide du XX siècle, la République française redonnait symboliquement au génocide arménien une place dans la mémoire collective de l'humanité. si cette reconnaissance a pu être considérée comme un achèvement pour certains, nous devons désormais aller plus loin, pour éviter toute concurrence des mémoires et toute inégalité de traitement entre les victimes et leurs descendants. La République se doit en effet de protéger l'ensemble de ses ressortissants. Nombre de descendants du génocide arménien ont trouvé refuge en France et sont Français. Face au négationnisme, y compris d'État, dont ceux-ci sont victimes, on doit s'en remettre non pas à l'arbitraire communautaire, mais bien à la justice de la République, pour garantir leur protection. C'est pourquoi il faut rechercher les outils juridiques les plus adaptés permettant de donner toute sa portée à la reconnaissance du génocide arménien et, plus largement, de réprimer la négation de l'ensemble des crimes de génocide et des crimes contre l'humanité, dans le strict respect des exigences constitutionnelles et conventionnelles.

À cet égard, il convient d'apporter la plus grande attention aux atteintes aux valeurs de la République que représentent les tentatives d'entrave numérique à l'interruption volontaire de grossesse. Nous visons spécifiquement les sites soupçonnés de pratiquer une désinformation sur l'avortement, sous couvert d'une approche neutre. Les conseils et informations dispensés aboutissent à ce que des femmes en recherche d'informations reçoivent des présentations biaisées, qui peuvent conduire à reporter ou mettre en doute leur souhait d'avorter. Les conséquences humaines pour la santé de la femme sont trop graves pour laisser faire. En 2017, la majorité précédente avait décidé d'instaurer un délit d'entrave numérique contre les sites dispensant ces informations, mais, dans la pratique, les associations de défense des droits des femmes nous alertent sur la persistance des entraves à l'IVG permises par les brèches de l'édifice législatif et l'interprétation restrictive qu'en fait le Conseil constitutionnel. Ainsi, aucun site de ce type n'a pu être condamné depuis la création de ce délit d'entrave numérique. C'est un sujet sur lequel il conviendra peut-être par un autre véhicule législatif. En attendant, il nous semble opportun de réaffirmer, dans le cadre de cet article, la nécessité de garantir le libre choix des personnes à disposer de leur corps et de viser l'article L. 2223-2 du code de la santé publique, afin que les nouvelles dispositions de l'article 19 soient applicables aux contenus entrant dans le cadre du délit d'entrave numérique à l'IVG.

: La parole est à M. Claude Malhuret. Mes chers collègues, les réseaux sociaux sont devenus dangereux ; ils injurient, ils humilient, ils blessent, et parfois pire. Ils commencent à miner la démocratie. le législateur, ici même, à l'Assemblée nationale, au Parlement européen ou au Congrès américain, a tenté d'y mettre un peu d'ordre. Pour l'heure, nous avons en grande partie échoué.

puisqu'elles portent sur la modération et qu'aucun juge ne pourra jamais intervenir efficacement sur les millions de messages postés quotidiens sur les réseaux sociaux- c'est exactement ce que vous avez dit il y a un instant, monsieur le secrétaire La raison de notre impuissance, c'est que nous avons cédé à l'argumentaire des plateformes numériques et de leurs milliers de lobbyistes, expliquant qu'ils étaient de simples hébergeurs des messages émis par leurs abonnés et non, comme la presse, des éditeurs responsables des contenus. Ce raisonnement les exonère de la responsabilité des contenus illicites, mais c'est évidemment une fiction : en effet, ces plateformes ne se contentent pas d'héberger des contenus. Leur est même à l'opposé, aboutit, par l'intermédiaire des algorithmes, à sélectionner les contenus les plus discutables, les plus polémiques, les plus violents- ce sont ceux qui génèrent le plus d'émotion, donc le plus de messages et le plus de fric. Certains disent, en parlant de la modération, que l'on ne peut confier la censure aux plateformes et que nous devons la réserver au juge. Bien sûr, mais c'est dès aujourd'hui que la censure est confiée aux plateformes, qui plus est en amont, puisque c'est par l'usage de ces algorithmes que les plateformes suppriment ou dégradent la visibilité des contenus, disons, normaux, au profit des plus dangereux. Loin d'être de simples hébergeurs, ces plateformes sont donc bien, par la sélection qu'elles opèrent dans la présentation, des producteurs de contenus ; elles doivent en assumer la responsabilité, comme, par exemple, les éditeurs de journaux qui sont responsables de leurs articles et des courriers des lecteurs qu'ils sélectionnent. C'est le sens de cet amendement, qui vise à maintenir le régime exonératoire de responsabilité pour les sites dont l'activité n'excède pas celle d'un simple hébergeur et à rendre enfin responsables les autres sites pour les contenus qu'ils diffusent, bien entendu Quel est l'avis de la commission ? cet amendement est contraire au droit européen actuel, puisqu'il tend à ajouter des critères plus restrictifs que la définition posée par la directive dite « e-commerce » et par la Cour de justice de l'Union européenne. il exclurait du statut d'hébergeur des plateformes actuellement protégées par le droit européen, dont la loi pour la confiance dans l'économie numérique n'a pu qu'assurer la transposition fidèle.

de supprimer non seulement les contenus, mais aussi le compte lui-même du président des États-Unis. Certains y ont vu une mesure liberticide, qui bridait la fonction même des réseaux sociaux

au renversement en direct des principes de la République américaine. Souvenez-vous de ces gens qui sont entrés dans le Capitole pour assassiner nos collègues sénateurs

pour que la mesure soit équilibrée et pas seulement contraignante pour les utilisateurs, je vous propose également un dispositif législatif visant à interdire les entraves à la liberté d'expression sur les réseaux sociaux par les géants du numérique. numérique. L'amendement que notre assemblée a l'honneur d'examiner vise à interdire la censure de propos licites et non punis par la loi française sur ces réseaux et à mettre en place une voie de recours spécifique, rapide et dématérialisée, en vue de permettre aux utilisateurs entravés de contester les mesures prises par les réseaux sociaux. Les entraves à la liberté d'expression par les géants d'internet, propriétaires des réseaux, sont devenues monnaie courante et présentent de vrais problèmes démocratiques, notamment quand il s'agit de censurer les publications de parlementaires ou d'autres élus, d'autant que cette mesure concerne toujours, ou presque, le même sujet : la critique de l'immigration et de l'islamisme. À la fin du mois de janvier, le compte Twitter de notre collègue Sébastien Meurant a ainsi été suspendu pour avoir diffusé la photo d'une femme en burqa et rappelé la loi. doit s'armer et s'affirmer au fil de la transition numérique et assurer les conditions de la liberté d'expression. Les problèmes de notre société ne se régleront pas en mettant un modérateur, aussi omnipotent soit-il, sur un réseau social, réseau qui n'est qu'une fenêtre d'expression, souvent révélatrice de malaises profonds du quotidien de nos compatriotes. C'est faux ! Les réseaux sociaux sont devenus de vrais médias d'opinion et d'information que la loi doit réguler, pour y assurer l'égalité de traitement et la sécurité de la liberté d'expression, comme ailleurs dans la société. Les 26 et 27 mars dernier, les comptes Twitter de Marika Bret, figure de, et de la vice-présidente d'une association pro-laïcité ont été suspendus pour avoir posté la une du journal satirique représentant Erdogan dénudé. Certes, ce n'était pas d'une grande finesse, avouons-le, mais ces méthodes de censeurs sont inacceptables. Le sultan turc n'aurait pas fait mieux

Quel est l'avis de la commission ?

Il est seulement prévu par la loi pour la confiance dans l'économie numérique que le signalement abusif aux hébergeurs d'un contenu en vue d'en obtenir le retrait peut être sanctionné pénalement, mais la plainte ne vise pas tant la plateforme qu'un autre utilisateur du réseau. Par cet amendement, il s'agit donc de créer un nouveau délit, sanctionnant la suppression par une plateforme d'un contenu dont l'illicéité n'est pas manifeste.

des censures directes de la part des plateformes pour éviter de courir ce risque. Par ailleurs, je me dois de rappeler qu'une plateforme n'est pas un service public, donc les responsables doivent pouvoir continuer à à y modérer des contenus publiés. Ces derniers, bien que parfaitement licites au regard du droit pénal, ne sont pas autorisés par leurs règles générales d'utilisation. En outre, les peines proposées sont calquées sur celles qui étaient prévues par la loi Avia, déjà jugée

Il est important qu'une approche transversale soit adoptée au niveau de l'Union européenne concernant la régulation des services numériques, une approche permettant de préserver les droits et libertés fondamentaux des utilisateurs de ces services. C'est une bonne chose que la France occupe sa place dans ce débat européen, mais je regrette que la question du respect des droits fondamentaux en matière numérique, qui appelle un grand débat démocratique, soit abordée seulement en urgence et de manière marginale, dans une loi dont ce n'est pas l'objet.

des mesures qui ne sont qu'une reprise d'un projet de texte n'ayant pas encore été discuté au Parlement européen, au risque que nous devions légiférer de nouveau sur le même sujet dès que le texte européen sera adopté. Il y a un temps pour tout : les transpositions européennes doivent être réalisées après leur discussion et leur vote, et pas avant ! Une fois encore, le Gouvernement se précipite et ne permet pas de créer les conditions d'un débat au niveau national sur ce sujet de société. Plus généralement, les mécanismes concourant à la propagation des contenus haineux, ainsi que les instruments qui viseraient à les réguler, ne sont pas suffisamment pris en compte pour une lutte efficace contre la haine en ligne. De plus, comme dans le reste de cette loi, il y a beaucoup le déclaratif : des moyens qui seront réellement mis en place par les plateformes ? Les amendes en cas de non-respect de ces nouvelles obligations seront-elles suffisantes pour que les plateformes respectent ces nouvelles contraintes ?

du 24 juin 2020 visant à lutter contre les contenus haineux sur internet, dite « loi Avia nul besoin de rappeler que cette loi a fait l'objet de nombreuses censures de la part du Conseil constitutionnel. Si les dispositions de cet article visent essentiellement à renforcer les pouvoirs de sanction du Conseil supérieur de l'audiovisuel, les auteurs de cet amendement estiment, d'une part, qu'elles n'ont pas leur place dans ce texte, et, d'autre part, qu'elles portent atteinte à la liberté d'expression. Ne nous trompons pas de combat : internet est un espace de liberté d'expression de ses convictions, de communication de l'information et de critique de l'action des pouvoirs publics. Il est Il est difficile de comprendre en quoi la lutte conte les prétendus séparatismes devrait y être menée. Pour ces raisons, le groupe Écologiste-Solidarité et Territoires demande la suppression de ces dispositions. Quel

Quel est l'avis du Gouvernement ? Je ne reviens pas sur l'argumentaire que j'ai déroulé sur l'avis du Conseil constitutionnel. Ce dernier ne me paraît pas applicable en l'espèce, puisque le Conseil ne s'est jamais prononcé au fond sur les éléments qui sont évoqués.

obligation de retrait ou blocage dans les vingt-quatre heures, mais à titre provisoire, et validation par un juge statuant en référé. À l'époque, nous n'avions pas convaincu, mais le Conseil constitutionnel est passé par là, et, pour tout dire, je ne sais plus, je le confesse, si ce motif a été précisément examiné. En tout cas, nous y voilà de nouveau : nous proposons de combiner l'urgence du retrait et l'intervention du juge, qui est le seul garant de la protection des libertés publiques.

CSA. Cette exclusion est partiellement bienvenue et justifiée. On comprend certaines des raisons qui ont poussé la commission à aller en ce sens. Plusieurs des obligations introduites n'ont pas vocation à s'appliquer aux moteurs de recherche, puisque ceux-ci ne donnent pas accès à des contenus mis en ligne par leurs propres utilisateurs, qui sont des personnes qui procèdent à des recherches de sites internet. Effectivement, les obligations tenant aux conditions générales d'utilisation du service, à la notification de contenus, au traitement de ces notifications, aux mécanismes de recours des utilisateurs contre les décisions prises par les plateformes, ou encore à l'utilisation abusive du service, n'ont pas lieu de s'appliquer aux moteurs de recherche. Nous voulons bien en convenir. En revanche, eu égard au rôle que jouent les grands moteurs de recherche dans l'accès aux contenus en ligne et à la responsabilité qui en découle, nous pensons qu'il faut leur appliquer tout de même plusieurs des obligations qui visent les plateformes en ligne. Il s'agit surtout des obligations les plus importantes, notamment l'évaluation par ces plateformes des risques systémiques liés à leur service et l'adoption de mesures d'atténuation de ces risques sous le contrôle du régulateur. Elles permettront la mise en place par les moteurs de recherche de mesures de lutte contre les contenus illicites, par exemple par l'adaptation de leur algorithme de classement, pour rétrograder de façon systématique ce type de contenu et limiter drastiquement leur visibilité.

Assouline. Conformément à la position qu'il a prise à l'occasion de l'examen de la proposition de loi visant à lutter contre les contenus haineux sur internet, le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain souhaite introduire les moteurs de recherche dans le champ de la régulation du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

S'il est vrai que les réseaux sociaux constituent les principaux vecteurs d'échanges de propos haineux illicites, nous estimons que cette justification ne suffit pas à retirer les moteurs de recherche du champ de la régulation du CSA.

La mise en oeuvre de droits de recours prévus par l'article 19 au bénéfice des personnes qui voient leurs contenus supprimés par les plateformes ne va pas assez loin. Permettre uniquement un recours en interne auprès de la plateforme est insuffisant. Seule l'autorité judiciaire devrait évaluer au cas par cas les recours formés par les utilisateurs contre les opérations de modération. Il est important de s'appuyer sur les juges pour toute décision de ce genre. Après l'échec cuisant de la loi Avia,

Les citoyens français ont des devoirs, mais également des droits, et la censure est une pente dangereuse. Choisir le juge comme arbitre est judicieux pour éviter des décisions liberticides. C'est la raison pour laquelle nous proposons d'instaurer une obligation de retrait ou de blocage en vingt-quatre heures, à titre provisoire, d'un contenu haineux notifié qui serait manifestement illicite, jusqu'à la validation par le tribunal judiciaire statuant en référé.

notifié, avec une sorte de référé confirmation. Les contenus en cause devraient être retirés temporairement par tout intermédiaire technique, qui ferait valider sa décision par le juge des référés.

L'amendement n° 436 vise à réserver à l'autorité judiciaire l'examen du recours formé par les utilisateurs contre des décisions de modération.

tend à créer un délit de non-retrait en vingt-quatre heures de certains contenus illicites par les opérateurs de plateforme en ligne. C'est très exactement ce qui a été censuré par le Conseil constitutionnel dans la loi Avia. De plus, prévoir un délai couperet de

du Conseil supérieur de l'audiovisuel, ce qui est contraire à la position du Sénat. La nouvelle régulation des plateformes, qui sera valable à peine deux ans, doit se concentrer sur les réseaux sociaux à fort trafic, principaux vecteurs d'échanges de propos haineux illicites. En effet, les moteurs de recherche, dans leur fonctionnement technique, leur finalité et leurs conséquences sur la viralité d'un contenu se distinguent substantiellement des réseaux sociaux, puisqu'ils n'hébergent pas, mais dirigent vers. On ne peut donc leur appliquer le même régime.

Or, vous le savez, tôt ou tard, et le plus tôt sera le mieux, il faudra revenir à des dispositions de ce type. Pourquoi ?

n'est pas exorbitant. C'est la seule manière de protéger la personne. Par ailleurs, le fait que la décision de retrait ou de non-retrait soit prise par un juge judiciaire constitue une garantie absolue. On voit bien ce qu'ont donné les dispositifs consistant à demander aux différents organismes éditeurs, auteurs et porteurs d'effectuer une censure des messages haineux. Cela a abouti à des choses parfaitement arbitraires, aléatoires. J'y insiste, seul le juge est ici pertinent. il faut aller vite ; deuxièmement, il faut donc donner à la personne la possibilité d'obtenir la suspension dans des délais rapides la décision de retrait éventuel ne peut pas être prise par l'organisme ou par la société. Elle doit être prise par un juge. C'est la raison pour laquelle il existe des procédures en référé. Je veux bien que l'on nous dise que c'est matériellement difficile à mettre en oeuvre,

provenant de certaines entités publiques, telles que Pharos, ou d'associations de lutte contre la haine en ligne. Toutefois, la rédaction de la commission impose aux signaleurs de confiance un critère général d'indépendance. Or les tiers de confiance sont un phénomène récent. En pratique, leur organisation est très variable et peut reposer en partie sur des financements extérieurs. Il paraît donc préférable, afin de garantir le caractère opérant du dispositif utilement introduit par la commission des lois,

l'avis de la commission ?

les mesures radicales de suspension ou résiliation du compte d'un utilisateur, ou de suspension de l'accès au dispositif de notification, ne peuvent être prises dans l'urgence et unilatéralement par une plateforme que de manière provisoire. Le dispositif de recours reposant sur une procédure interne est insuffisant sans le contrôle de l'autorité judiciaire. Tout comme pour le retrait ou le blocage, cet amendement a donc pour objet d'appliquer dans de tels cas ce principe élémentaire, afin d'écarter tout risque de suspension ou de résiliation abusive. Les plateformes ont déjà un pouvoir important ; il est nécessaire que l'autorité judiciaire puisse contrôler les suspensions ou fermetures de comptes avant une décision définitive, afin d'éviter les abus et les phénomènes de censure par

amendements visent, comme les précédents, à réintroduire le juge dans le processus de retrait des contenus haineux.

retirés en cas de contre-notification par leur auteur, à charge pour le notifiant de saisir le juge des référés. Cela peut poser des problèmes relatifs à l'intérêt à agir du requérant : une notification de contenu haineux illicite peut être adressée à un hébergeur par toute personne, sans qu'elle ait à justifier d'être personnellement lésée par ledit contenu, alors que son action devant le juge devra bien s'appuyer sur un tel intérêt, sauf à permettre une sorte d'action populaire.

et lui donner tort, alors même que la plateforme engage sa responsabilité pénale et civile si elle ne retire pas promptement ces contenus. Si l'amendement n° 437 était retenu, la plateforme ne pourrait suspendre ou résilier le compte d'un utilisateur que de manière provisoire, à charge pour elle de saisir le juge des référés.

et conduirait à un contrôle plus restreint des outils des plateformes. La formule « en matière de » a une visée plus favorable que celle que vous proposez. Il convient donc, selon le Gouvernement, de conserver une disposition large, de manière à s'assurer que les plateformes conduisent l'évaluation de leurs outils la plus complète possible.

L'article 19 prévoit que les plateformes permettent au CSA d'avoir accès aux principes de fonctionnement des outils automatisés auxquels ils ont recours pour répondre à leurs nouvelles obligations, ainsi qu'aux paramètres utilisés par ces outils. La question de la transparence des algorithmes est posée.

Cet amendement est une réponse. On demande aux Gafam non pas de remettre ces informations au premier venu, mais de les confier à une instance de régulation chargée de les vérifier. Si ce n'est pas fait, nous ne pourrons pas contrôler la pertinence de ces outils ; même le CSA ne le pourra pas. L'obligation de transparence proposée dans l'article 19 est incomplète. Une fois de plus, ce projet de loi affiche des intentions ou des principes, mais cela ne suffit pas. Il est crucial de pouvoir juger sur pièces, c'est-à-dire de pouvoir contrôler la conformité des algorithmes aux principes d'un espace public démocratique.

Il convient donc de prévoir dans la loi un accès direct aux algorithmes. J'aimerais également évoquer la question des moyens humains dont le CSA a besoin pour accomplir au mieux sa nouvelle mission de contrôle des plateformes. Il lui faudra le financement nécessaire afin de débaucher, des ingénieurs qualifiés pour ce travail, sachant que les meilleurs d'entre eux se vendent à prix d'or et que les plateformes disposent de moyens quasi illimités. Dans tous les cas, la question

la capacité de régulation du CSA par collecte automatisée des données. Dans la mesure où l'on veut lui confier un rôle de régulateur, il ne faut pas trop restreindre ce rôle. Si l'on tire

ou après inscription sur le site en cause ». Or de nombreux acteurs visés par le champ du dispositif ne présentent rien sur l'internet ouvert,

faire l'objet de contrôles. Afin de ne pas limiter le caractère opérationnel de la régulation, nous proposons de préciser ce que sont les données publiques accessibles par le CSA dans le cadre de sa collecte automatisée, en expliquant qu'elles comprennent bien celles des sites qui nécessitent la connexion à un compte. Quel

M. Stéphane Artano. Cet amendement a pour objet les sanctions pécuniaires dont sont passibles les opérateurs de plateformes en ligne en cas de manquement à leurs obligations. S'il est nécessaire de prévoir des sanctions à l'encontre des opérateurs qui ne se conformeraient pas aux mises en demeure du CSA, en revanche pas possible d'admettre qu'ils puissent être exonérés de sanctions pécuniaires dans le cas où un autre pays les aurait déjà condamnés pour un même manquement. Une sanction de ce type doit être rendue souverainement, sans qu'il faille rechercher si, à l'étranger, une administration ou une juridiction aurait également sanctionné l'opérateur, d'autant que les seuils proposés nous paraissent relativement insuffisants au regard des bénéfices que dégagent ces plateformes numériques.

risquerait d'entraîner une disproportion dans les sanctions.

sont applicables pour les auteurs présumés de provocations à la haine et de délits de provocation prévus à l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881. Selon le Conseil national des barreaux, user des procédures rapides de jugement dans le cadre de ces délits revient à méconnaître la technicité de ces dossiers et les garanties procédurales de la loi de 1881. Les infractions de provocation à la haine, notamment en ligne, requièrent une expertise de la part des enquêteurs. Les magistrats rencontrent également plus de difficultés à matérialiser des faits de cyberharcèlement et à qualifier pénalement les infractions du champ virtuel. Dans la pratique, ce type de contentieux se heurte à un manque de personnel formé au sein des services enquêteurs. L'exploitation du matériel informatique et les investigations techniques sont confiées à des experts privés. Ce manque de moyens allonge considérablement les délais d'analyse des données recueillies. Nous partageons donc le constat que la procédure de comparution immédiate, qui présente un caractère expéditif, n'est pas adéquate pour juger ce type d'infractions. Enfin, il convient de ne pas nier la spécificité et le caractère sensible des délits mentionnés par la loi du 29 juillet 1881, repose sur un équilibre entre la liberté d'expression, la liberté d'opinion et les abus commis. La France, pays très attaché à la liberté d'expression, doit maintenir un cadre spécifique pour ce type de contentieux. Pour l'ensemble de ces raisons, le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires demande

dans un système qui met totalement à la poubelle le principe même de protection de ceux qui sont soumis à la loi du 29 juillet 1881. C'est très grave ! Cela l'est déjà dans les circonstances

Son absence est un dur silence pour nous. Nous comprenons bien que, finalement, ce qui est touché par ce texte est la loi sur la liberté

identiques de suppression. Cet article permet la répression rapide, par la comparution immédiate, des responsables des infractions les plus graves prévues par la loi de 1881 lorsqu'ils agissent comme des individus seuls responsables de leurs actes. Il n'exclut pas les

Comme vous êtes attachée au droit, vous savez que, constitutionnellement, n'importe quel ministre est habilité à représenter le Gouvernement. Il fait partie du jeu politique que l'opposition dénonce l'absence de tel ou tel. Quand cette même opposition est au pouvoir comme vous l'avez été, elle ne le fait pas-

En d'autres termes, le journaliste qui s'exprime en son nom, et non pas comme complice de son directeur de la publication, serait inclus dans le champ de cet article. C'est très dangereux.

vise justement à éviter l'application de procédures de jugement rapide dans tous les cas où un organe de presse est concerné.

qui n'est pas concerné par cette dérogation à la non-application de la comparution immédiate : les journalistes qui s'expriment sous leur nom sur les réseaux sociaux, les lanceurs d'alerte-

Ce fait est suffisamment important pour que je le souligne. Ce n'est pas à moi, à titre personnel, qu'il a ainsi été porté atteinte. C'est à la présidence, à la sérénité de son exercice et à une règle essentielle dans l'exercice de la présidence